monsieur le président

Parmi les nombreuses solutions possibles, il apparaît essentiel que le statut de lanceur d'alerte puisse leur être octroyé afin de mieux les protéger. Cette possibilité permettrait de mieux prévenir les dérives pouvant être observées dans les services publics ou dans les associations et les fondations qui ont, par exemple, signé un contrat d'engagement républicain. Aussi, une telle possibilité doit être expressément indiquée dans la loi afin d'éviter que les personnes constatant ces atteintes ne soient exposées aux représailles de ceux qui porteraient atteinte aux principes républicains. est l'avis de la commission ? Le statut de lanceur d'alerte est conféré aux personnes qui signalent un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. Il semble disproportionné de l'étendre aux signalements de manquements au contrat d'engagement républicain, qui ne constituent d'ailleurs pas forcément des infractions pénales. L'avis de la commission

vise à faire cesser le versement de subventions municipales à des associations dites « loi 1901 » qui exerceraient une activité ne respectant pas les valeurs constituant le socle de notre pacte républicain. Je pense aux exigences minimales de la vie en société, telles que le respect de la dignité, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, le respect du droit ou encore la condamnation de tout discours de haine à l'encontre de toute personne ou tout groupe de personnes. De telles subventions ne peuvent être acceptées. Pour cela, il faut demander aux maires, représentants de la puissance publique au coeur de la vie quotidienne de nos concitoyens, de mettre fin à tous les avantages ou subventions quels qu'ils soient et d'en exiger la restitution, à défaut de quoi de lourdes sanctions dissuasives devront être prononcées. prononcées. Je rappelle que la mairie de Strasbourg a pris la décision de subventionner la construction de la mosquée Eyyûb Sultan à hauteur de 2,5 millions d'euros. Madame la ministre, je vous ai entendue à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas besoin de mémo pour savoir que l'organisation turque Millî Görüs est particulièrement curieuse. Je partage vos propos nous ne pouvons cautionner que la mairie verte de Strasbourg subventionne une mosquée soutenue par une association qui ne condamne ni l'islam politique ni l'apostasie. Je rappelle que l'organisation Millî Görüs (CIMG) a été créée à la fin des années 1960 en Allemagne par Necmettin Erbakan, ancien Premier ministre turc, et s'est installée progressivement en Europe occidentale, sous l'impulsion de membres de la diaspora turque présente outre-Rhin. La CIMG est aujourd'hui présente dans soixante-dix lieux de culte en France. Un autre groupe turc, le Comité de coordination des musulmans turcs de France, pilote 270 des quelque 2 500 mosquées présentes sur le territoire. Ainsi, 14 % des mosquées de notre pays sont liées à la Turquie. Je voudrais vous citer Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble- une ville malheureusement célèbre ces derniers temps pour des événements peu républicains -et spécialiste de la Turquie contemporaine, qui revenait sur les motivations du groupe : « Ils ont le même projet que les Frères musulmans : faire de l'islam politique.

pas forcément opportun. En outre, punir d'un an de prison la non-restitution de la subvention dans les trois mois semble disproportionné. Le droit en vigueur punit déjà du délit d'abus de confiance

un soutien clair aux maires et à la libre administration des communes en leur permettant de refuser, en cas de soupçons de radicalisme, de mettre à disposition d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une association un local communal. Aujourd'hui, les pouvoirs du maire sont limités par le principe d'égalité et la liberté de réunion. Il ne peut empêcher une réunion communautariste qui ne menace pas clairement l'ordre public. Cet amendement affirme au contraire que, par sa fonction, le maire peut réunir un faisceau d'indices suffisant pour refuser la mise à disposition d'un local communal en cas de soupçons de radicalisme. Le maire dispose d'une place primordiale, à portée des coups à prendre, mais également à portée des coups à donner. La loi doit lui permettre d'empêcher concrètement la propagation conquérante des idéologies islamistes dans les limites de sa commune. Vous êtes nombreux à avoir été élus locaux, mes chers collègues, et à savoir combien cette problématique est prégnante. Je vous invite par conséquent à voter cet amendement pragmatique pour lutter contre l'islamisme, redonnant toute sa place à la subsidiarité.

permet déjà aux maires de fixer par règlement intérieur les conditions d'usage des locaux compte tenu de la nécessité du maintien de l'ordre public. Laissons donc les collectivités gérer. L'avis de la commission

Il s'agit d'interdire le fait qu'une commune permette par la location, le prêt à titre gracieux, voire le bail emphytéotique qu'une salle municipale devienne un lieu de culte. Il n'est question ni de temps ni de lieu, mais véritablement de principe : une collectivité locale ne doit en aucun cas se détacher de la neutralité dans ses rapports avec les cultes.

En effet, le seul motif d'atteinte à l'ordre public et de menaces en la matière ne saurait suffire. Même si un règlement d'occupation des salles peut être porté par le maire, il convient d'inscrire cette possibilité dans la loi,

165 rectifié. Pour nous, la décision d'autoriser l'utilisation de salles municipales et la détermination des conditions dans lesquelles cela s'effectue appartiennent au maire, qui dispose de la compétence exclusive

Les conditions financières de la mise à disposition au bénéfice d'un culte ne doivent pas conduire à caractériser une libéralité, en raison de la prohibition par l'article 2 de la loi de 1905, que chacun ici connaît.

le service civique mobilise annuellement un nombre de jeunes de plus en plus important. En 2021, le dispositif doit permettre à 245 000 jeunes de s'engager dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Il offre à toute personne volontaire l'occasion de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général. Au regard des objectifs assignés aux dispositifs et du nombre de jeunes engagés dans ce cadre, les organismes agréés au titre du service civique se doivent de respecter les valeurs de la République.

Les conséquences tirées du non-respect de ce contrat, c'est-à-dire le retrait de l'agrément, seront fixées par voie réglementaire. La majorité des jeunes qui s'engagent en mission de service civique sont accueillis par des organismes sans but lucratif. Ceux-ci bénéficient d'un aide pour l'accompagnement des jeunes pendant leur mission, mais également d'une aide destinée à financer la formation civique et citoyenne des jeunes. Notre amendement vise donc à ce que ces aides, dans le respect du principe du contradictoire, soient restituées par l'organisme sans but lucratif n'ayant pas respecté le contrat d'engagement républicain

Naturellement, les gouvernements cherchent comment combattre et endiguer un tel phénomène. Ce projet de loi pourra indéniablement apporter des réponses et des solutions. Par cet amendement, nous cherchons à ouvrir une nouvelle voie, celle de la création d'une qualification juridique de « comportement sectaire qui serait répréhensible. En effet, les notions de « secte » et de « comportement sectaire » permettraient d'isoler et de réprimer certaines pratiques extrémistes, tout en les distinguant des pratiques religieuses, qui, le plus souvent, ne posent pas de problème et demeurent pacifiques et respectueuses de l'ordre républicain. L'introduction d'une telle qualification pénale permettrait donc de condamner certains courants

comme je l'ai exposé longuement hier. Nous avons lancé un certain nombre d'actions, notamment la mise en place d'un conseil d'orientation de la lutte contre les dérives sectaires. Reste que, à ce stade, il n'y a pas de définition juridique de la secte, pas plus qu'il n'y a de définition juridique de la religion. Le législateur est respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de la laïcité. Dans tous les débats, nous avons toujours refusé de définir dans la loi ce que serait une religion ou une secte, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion, de religion, qui sont garanties par les différents textes fondamentaux. Je voudrais tout de même rappeler que la lutte contre les dérives sectaires est une priorité de notre action. Celles-ci sont réprimées par l'article 223-15-2 qui sanctionne de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse [ ...] d'une personne en état de sujétion psychologique

Christian Estrosi, maire de Nice, considérer qu'un imam islamiste est un relais social important. Imaginons Samia Ghali, ancienne collègue et toujours troisième adjointe à la mairie de Marseille, se rendre aux grands événements organisés par une mosquée qui diffuse des textes appelant au djihad et au meurtre des apostats. la maire de Strasbourg vouloir subventionner une mosquée islamiste affiliée au pouvoir du dictateur Erdogan. Effrayant, non ? Pourtant, toutes ces histoires sont vraies et très récentes ! La liste, notamment à Marseille, n'est pas exhaustive, mais, par charité chrétienne, par charité chrétienne, par charité républicaine et par rondeur sénatoriale, comme dirait l'ancien maire de Marseille et vice-président du Sénat, je m'arrête là. Vous seriez tous d'accord, mes chers collègues, pour dénoncer ces agissements moralement et politiquement condamnables. Et vous auriez raison ! Mais cela ne va pas assez loin : année après année, les mêmes cas se répètent. Ces idiots utiles, qui ressemblent à s'y méprendre

Non seulement ce système affaiblit notre démocratie, mais il légitime et renforce les islamistes dans les quartiers. Il faut purger notre système politique de tous ceux qui alimentent ce système et laissent pourrir la République Refuser cet amendement n'aurait qu'une seule signification : faire de vous, à votre tour, des complices, certes indirects, mais complices quand même, de ce système islamo-clientéliste ! Le temps ! Mes chers collègues,

posséder un budget d'un certain montant et agir sur le plan national. Par ailleurs, ces associations et fondations sont déjà régies par un ensemble de contrats préexistants, qu'elles doivent notamment signer au moment de l'obtention d'une subvention. fait que la signature d'un contrat d'engagement républicain conditionne la reconnaissance de l'utilité publique d'une association ou d'une fondation.

par l'État d'un agrément aux associations loi 1901 et aux associations régies par le droit d'Alsace-Moselle et à la reconnaissance d'utilité publique des associations et fondations le respect de la charte des engagements réciproques- nous l'avons déjà évoquée -, et non celui des principes du contrat d'engagement républicain.

l'inutilité d'une telle mesure au regard du cadre juridique actuel, mais je voudrais insister sur un point. Le Gouvernement et la majorité souhaitent qu'aucun denier public ne soit attribué à des associations antirépublicaines. Cet objectif me semble faire consensus parmi nous. Toutefois, n'est-ce pas au final juste reporter le problème ? Ces associations ou groupements de fait trouveront leur financement ailleurs, notamment par le biais de dons probablement non déclarés. Là, ils passeront directement sous les radars de la puissance publique. En d'autres termes, au lieu de nous donner les moyens de lutter contre des phénomènes effectivement dangereux, nous allons laisser le soin aux élus locaux d'identifier et de gérer des problèmes qui pourront se faire jour chez eux. D'ailleurs, avons-nous ne serait-ce qu'une estimation des associations visées qui perçoivent ces subventions ?

importants. Or les associations doivent se mettre en conformité avec le tronc commun d'agrément qui est complété par le projet de loi au plus tard le 9 mai 2022, en application du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017. En matière sportive, le choix est fait d'encadrer l'application dans le temps de manière plus longue, compte tenu des jeux Olympiques de 2024, notamment. Pour les autres associations agréées par l'État de jeunesse et d'éducation populaire, qui sont un grand nombre, il nous semble indispensable de pouvoir redéfinir avec précision la mise en oeuvre de l'article 7 plutôt que de dépendre d'un décret d'application ancien. En outre, l'article 7 implique un nouveau système d'information pour la gestion interministérielle des agréments, afin que l'État et l'ensemble des autorités administratives intéressées puissent à la fois enregistrer et avoir accès à l'information sur la souscription du contrat d'engagement républicain. Une modification importante du compte association est dès lors indispensable. Les associations, fédérations et unions qui n'auront pas adressé une nouvelle demande d'agrément avant la fin du délai légal ne pourront plus prétendre au bénéfice de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire, ni du tronc commun d'agrément et, par voie de conséquence, notamment de subventions de l'État spécifiques. Il nous semble important d'encadrer dans le temps les décisions d'agrément pour en permettre la vérification dans le cadre du renouvellement de la décision. Ce délai doit être assez long pour ne pas entraver l'exercice de la liberté d'association, à laquelle le Gouvernement est très attaché, et apporter suffisamment de garanties d'exercice aux associations. En matière de jeunesse et d'éducation populaire, depuis la loi du 17 juillet 2001, aucune condition de durée n'était prévue. Cela complexifiait la gestion des agréments des associations, qui doivent par ailleurs toutes satisfaire aux conditions du tronc commun d'agrément, d'une durée de cinq ans. de cinq ans. Comme cela est déjà prévu pour les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, l'uniformisation des durées sur cinq ans entre l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire et le tronc commun d'agrément simplifierait la gestion pour les administrations chargées de cet agrément,

vie associative estime que la rédaction actuelle de cet article crée une présomption de responsabilité du fait d'autrui susceptible d'entraîner la dissolution d'une structure en raison du comportement de ses membres, ce qui va à l'encontre de l'article 121-2 du code pénal, qui dispose qu'une personne morale est responsable pénalement des seules infractions commises par ses organes ou représentants. Peut-on représentants. Peut-on légitimement estimer qu'une association a les moyens de contrôler l'action de ses membres ? Cette disposition crée une situation d'insécurité juridique pour les associations,

contraire à la Constitution en raison de son caractère disproportionné, qui empêche de protéger la liberté d'association en tant que principe fondamental reconnu par les lois de

dans le sens d'une présomption de responsabilité du fait d'autrui. Il est essentiel, dans tout notre édifice juridique,

Je n'aurais pas pris la parole si je n'avais pas un exemple précis en tête. J'ai en effet saisi depuis plusieurs mois maintenant les services du ministre de l'intérieur d'une demande de dissolution d'une association ouvertement raciste,

nos valeurs et nos principes républicains en substituant des lois religieuses aux lois de la République. Cet amendement vise à mettre un coup d'arrêt à ces ennemis

pourraient être dissous les associations ou groupements ayant pour but, sans que cela se manifeste nécessairement par la force, « d'attenter à la forme républicaine du Gouvernement ou aux principes de la démocratie ou de la souveraineté nationale ». Quel est l'avis de ? Cet amendement tend à modifier le motif de dissolution figurant au 3° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure afin de viser les associations qui se donnent pour objet d'attenter aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale, et non plus celles qui attentent par la force à la forme républicaine du Gouvernement. Je comprends votre intention, mon cher collègue, mais cette évolution ne me paraît pas souhaitable. Supprimer les mots « attenter par la force » risque de rendre la dissolution disproportionnée.

Nous ne ferons pas de procès d'intention, mais cette suppression nous interpelle. La société évolue, et nous nous devons d'accepter de faire évoluer les normes. Les questions de genre existent, et nous ne pouvons pas ostraciser plus encore certaines Françaises et certains Français au motif que les plus réfractaires d'entre nous voudraient éviter le débat sur ce sujet. Le présent amendement du groupe Écologiste- Solidarité et Territoires vise donc à rétablir l'alinéa 9 de l'article 8 dans sa rédaction initiale. Nous estimons en effet que la prise en compte de l'identité de genre est aussi importante que celle des autres motifs précités. Quel

législatif un peu trop permissif à l'égard de tels agissements qui encouragent la fracture de notre société. Cette affaire a mis en exergue la complexité des conditions de dissolution d'une association syndicale

vide juridique en donnant la possibilité au Gouvernement de prononcer la dissolution de toute association qui organise des réunions contraires aux principes fondamentaux que ce projet de loi entend conforter. L'interdiction explicite

aux principes républicains. Toutefois, d'un point de vue purement juridique, je rappelle en premier lieu que la protection constitutionnelle de la liberté d'association exige que la dissolution administrative d'une association ou d'un groupement de fait, dont les effets sont immédiats et définitifs, ne puisse reposer que sur des motifs

à raison de la couleur de peau, de l'origine ou de l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une religion pourrait être considérée comme propageant des idées tendant à encourager cette discrimination et tomber sous le

Je suis heureux, madame la ministre, que vous désapprouviez personnellement le comportement inacceptable d'un certain nombre de dirigeants de l'UNEF, et je ne partage pas l'avis de notre collègue, Mme Cohen, quant aux excuses rétrospectives qu'on avance maintenant pour justifier de tels comportements : le racisme à rebours ne vaut pas mieux que le racisme tout court

du code de la sécurité intérieure est applicable ou non pour sanctionner les dérives de l'UNEF ne me paraît pas tout à fait décisive. compte tenu de la position de fond que vous avez exprimée- je ne doute pas qu'elle exprime également celle de l'ensemble du Gouvernement -, si cet article était suffisant, j'imagine que vous auriez engagé la dissolution de l'UNEF. Cet

qui interdiraient à une personne ou un groupe de personnes d'y participer « à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée

ne déshonorerait personne dans cet hémicycle, bien au contraire. Je n'ai pas signé la demande de dissolution de l'UNEF, mais je suis en accord avec le président de mon groupe pour demander au minimum

Il a écrit ces mots : « C'était au début des années 2010, et, avec un ami blanc, on était allé à Paris à une réunion d'un collectif pour parler des discriminations que subissent les habitants des quartiers populaires. La réunion était ouverte à tous. À un moment, mon ami, blanc, a demandé à s'exprimer. Je ne sais plus trop exactement ce qu'il a dit, mais son intervention n'a pas plu aux organisateurs. Mon pote n'était pas un grand orateur, il n'avait pas l'habitude de parler en public, mais, en aucun cas, il n'avait été insultant. Au lieu de débattre avec lui sur le fond, l'un des responsables lui a dit : " Toi, t'es Blanc, t'es pas légitime pour venir ici et nous faire la morale ". Pourtant, mon poto avait grandi avec nous à la cité. C'était un frérot. Ses parents savaient à peine lire et écrire. Il avait quitté l'école à l'âge de 16 ans et, lui, était un vrai prolo. Il avait subi des discriminations sociales. J'ai dit à mon pote " Viens, on s'barre ", parce que j'ai vu qu'il commençait à être vénère. Et, en face, ça se voyait que ça ne se bagarrait pas. Mon pote avait été très blessé par cette remarque. Vraiment ! Et je me souviens de lui avoir dit

de fait dont l'objet ou l'action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et des personnes en situation de faiblesse, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l'ordre public et le respect de la liberté de conscience.

visant à réprimer la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous qui interviendrait sur le fondement d'une loi étrangère. Or il apparaît que la disposition est satisfaite par le droit pénal en vigueur lorsque l'on combine le principe de territorialité de la loi pénale et l'article 431-15 431-15 du code pénal, qui fait partie de la section du code pénal à laquelle renvoie précisément l'article L. 212-1 précité pour les modalités de répression de la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous. Au terme de ce principe, la reconstitution d'une association dissoute sur ce fondement pourra en effet être réputée commise sur le territoire français, dès lors que l'un des faits constitutifs aura lieu sur le territoire. Les mêmes peines seront en outre encourues. Nous proposons de supprimer la disposition introduite par la commission afin de ne pas complexifier l'articulation des dispositions en vigueur, qui la rendent superfétatoire. Quel

Ainsi, ce renforcement de la loi pénale nous paraît utile pour garantir la répression des associations ou groupements dissous en France, comme le CCIF, qui se reconstituent le lendemain de la publication du décret de dissolution sur le fondement d'une loi étrangère, réduisant à néant les efforts des pouvoirs publics.

il tue son voisin, doit-on dissoudre l'association et poursuivre ses membres ? Non, sans quoi plus personne ne s'inscrirait dans une association ou y partagerait des discussions avec les autres ! Ce projet de loi, n'exprimant pas son intention claire et initiale de vouloir lutter contre l'islamisme, perd la tête et en vient à amputer des libertés, droits et principes pourtant garantis à tous les citoyens. On ne peut étouffer les ennemis de la liberté avec des mesures législatives entravant les libertés de tous, sinon c'est déjà leur victoire. On touche ici du doigt les conséquences directes du refus de désigner et de cibler l'ennemi. Des citoyens et des associations vont se retrouver la cible de la loi, parce que celle-ci n'a pas voulu nommer et cibler précisément l'islamisme pour C'est pourquoi je demande aux membres de cette noble assemblée, qui ne partagent pas toujours mes idées, ce qui est étonnant, et ne sont pas tenus pour responsables de mes propos, de voter cet amendement et de refuser l'instauration d'un principe de responsabilité collective, étranger à l'esprit de notre droit.

pour présenter l'amendement n° 523. Une nouvelle fois, cet article pose un certain nombre de questions, notamment en matière de responsabilité des associations. Ainsi, le Gouvernement entend imputer plus clairement à une association les agissements de l'un de ses membres, tout en permettant de s'exonérer de la voie judiciaire pour procéder à une dissolution. dissolution. Il est vrai que, depuis la première version du texte, les parlementaires de la majorité et le Gouvernement ont mis de l'eau dans leur vin, le Conseil d'État lui-même considérant le texte initial comme méconnaissant sérieusement la liberté d'association. Il n'en demeure pas moins que tout cela reste difficilement compréhensible, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il est déjà possible de mettre en oeuvre juridiquement cette responsabilité collective. C'est ce qui ressort de la jurisprudence et des avis du Conseil d'État dans le cas de différents groupes ou associations : les Boulogne Boys en 2008, Envie de rêver en 2014 ou encore BarakaCity au mois de novembre dernier. La rédaction actuelle du texte tend à généraliser cette responsabilité collective ; pourtant, les dispositions actuelles sont amplement suffisantes.

un appel à la haine lancé sur Twitter par un individu se réclamant du Secours populaire ou de SOS Chrétiens d'Orient pourra-t-il engager la responsabilité de l'ensemble de l'organisation ?

Les risques qui pèsent sur la responsabilité des dirigeants bénévoles et qui conduisent à décourager la prise de fonction ont été pointés dans le cadre d'une proposition de loi relative à l'engagement associatif, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. de l'alinéa 15, couplée à celle de l'alinéa 20, fait peser ce même risque sur la prise de responsabilité bénévole, en ce que les dirigeants bénévoles deviennent responsables des agissements des membres de l'association, à condition qu'ils en aient été « informés Comment pourraient-ils prouver qu'ils n'avaient pas connaissance des agissements visés ? En outre, cette notion d'information, très floue, inflige une double peine pour le dirigeant bénévole, qui se trouve également dans une posture de dénonciation potentielle envers l'un des membres de son association.

pour contrôler les faits de leurs membres. Cet amendement vise à prévoir de n'imputer à l'association que les agissements de l'association elle-même ou ceux commis par ses dirigeants au nom de l'association.

la réduire. Ces modifications réduiraient l'efficacité opérationnelle du dispositif, alors que des garanties sont prévues pour assurer sa proportionnalité. Les agissements doivent avoir été réalisés en qualité de membre de l'association ou doivent liés à ses activités. Monsieur Ravier, je ne suis pas sûre que votre membre de l'association de boulistes, qui a tué son voisin, en tant que membre de l'association ou que son acte soit directement lié à son activité. Les dirigeants doivent avoir été informés des agissements individuels en cause et l'obligation de faire cesser les agissements reposant sur eux est une obligation de moyens, et non pas de résultat. Il nous semble que c'est relativement encadré

ces amendements. Les amendements n 347 et 348 de M. Meurant tendent à ajouter deux alinéas,

semblait justement que la période de trois mois permettait d'assurer ce fameux équilibre entre la liberté d'association et les contraintes qui pouvaient être imposées au travers d'une suspension.

par l'Assemblée nationale tendant à rendre renouvelable la mesure de suspension des activités d'une association ou d'un groupement de fait, dès lors qu'elle ou il fait l'objet d'une procédure de dissolution.

à l'instar de toute décision individuelle défavorable, en vertu du code des relations entre le public et l'administration. Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement souhaite rétablir cette possibilité de renouvellement de la mesure de suspension des activités d'une association. Je mets aux voix les amendements

C'est au contraire en assumant avec grandeur la République que nous voulons faire que nous les combattrons. Je voterai l'amendement, parce que je pense

de débattre, d'amender, de sous-amender en séance, parce que c'est notre droit constitutionnel de le faire. En travaillant dans des conditions satisfaisantes, ce soir, sur un sujet

sur les détails, à légiférer en commission, vont à contresens de ce que doit être le travail parlementaire. Évidemment, le groupe Union Centriste votera cet amendement, tout en rappelant, monsieur le président, messieurs les questeurs, mesdames, messieurs les présidents de groupe, à quel point le travail

de vote. Je pense que la République ne peut accepter aucune racialisation. Aucune ! Ni dans la société ni dans l'organisation publique. C'est une tentation qui est gravissime, et il faut évidemment, et clairement, réaffirmer qu'elle est contraire à nos principes communs. Je voterai donc cet amendement, je considère que l'exposé des motifs et les attaques, ou plutôt contre les organisations, me paraissent moins procéder de la volonté d'unir la Nation autour de ce refus de toute racialisation. Enfin, l'essentiel, c'est le texte de loi, et je l'approuve.

Je voudrais remercier le président Sueur, qui, par son intervention, a ramené cette partie de l'hémicycle à des traditions que nous avons en commun et qui sont républicaines. Il l'a rappelé avec force,

montre que nous avons bien la République en partage. On vient de la retrouver ensemble, après des moments un peu difficiles, mais, après tout, c'est la vie parlementaire. Je remercie enfin Stéphane Le Rudulier

concerne, j'ai un principe : l'universalisme républicain. Pour moi, la France, c'est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale,

Voilà deux ans, en novembre 2018, la Cour des comptes nous alertait sur le fait que les 900 millions d'euros de dépenses fiscales finançant les bonnes oeuvres des entreprises se trouvaient consentis en dépit de limites méthodologiques qui ne permettent pas de rendre compte du coût réel des mesures pour l'État. On ne sait ni vraiment ce que coûte à l'État la réduction d'impôt sur les sociétés de 60 % du montant du don ni quelle est l'efficience de la dépense fiscale et son potentiel de bénéfices pour l'intérêt général. général. L'intérêt général est en effet contestable pour bien des fonds de dotation, reconnaît une nouvelle fois la Cour. Cela s'explique par les critères, certes cumulatifs, mais très lâches, rendant possibles des abus, notamment sur la gestion des intéressés, même si, selon une étude 2016 par le cabinet EY, 40 % des répondants déclaraient une rémunération brute des dirigeants des fondations ou des fonds de dotation supérieure à 70 000 euros par an. Sans être désintéressée, cette rémunération ne dépasse pas trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 10 284 euros par mois. Le caractère extensif de la notion d'intérêt général est aggravé par le fait que l'État peine à assurer sa mission de surveillance et de contrôle. Les organismes bénéficiaires du mécénat n'ont pas à justifier d'une habilitation ou d'un agrément préalable de l'administration pour recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt, ce qui singularise la législation française en Europe. Comme le souligne la Cour, le mécénat est une niche fiscale qui demeure aussi fortement concentrée sur les très grandes entreprises, les vingt-quatre premières bénéficiaires de l'avantage fiscal représentant à elles seules près de la moitié du montant de la créance fiscale en 2016. Les dérives découlent également de la politique accommodante du Gouvernement, résumée par la vision de la secrétaire d'État chargée des associations, Sarah El Haïry, qui déclarait en 2019 qu'il qu'il fallait arrêter d'assimiler le mécénat d'entreprise a une niche fiscale, considérant que cette réduction d'impôt accordée aux fondations constituait non pas une dépense pour l'État, mais un investissement d'avenir.

9 ne comprend pour autant pas de mesures significatives. Pourtant, la dérive était prévisible dès la création de ce type de structure. Ces fonds de dotation sont des véritables niches fiscales. Ce régime est à questionner, puisque seulement 38 % des fonds

de la fraude fiscales.

Il détaille très précisément le montant des dégrèvements, des déductions d'impôt pour les dons, notamment ceux faits par les entreprises à des oeuvres ou des organismes d'intérêt général. Bref, il y en a deux pages et demie très détaillées, donc je ne vais pas passer la soirée là-dessus.

quand on est une structure, une entreprise, un particulier est extrêmement faible. Les chiffres sont disponibles. Aussi, je m'interroge très fortement sur l'intérêt et, surtout, sur la crédibilité de cette proposition. Voilà une dizaine de jours, M. Darmanin

Néanmoins, l'obligation de déclaration annuelle prévue par l'article 11 vise justement à concentrer les contrôles sur les entités les plus pertinentes, qui auraient particulièrement attiré l'attention des services fiscaux. Cela permettra d'avoir moins de contrôles, mais des contrôles ciblés.

toujours le cas dans le cadre de ce projet de loi. Cependant, je pense que nous avons tous été saisis par le monde associatif de ses inquiétudes au regard de procédures qui n'offrent pas

ainsi que le Haut Conseil à la vie associative, afin que les associations soient en mesure de faire valoir leurs droits lorsqu'elles sont en désaccord avec l'appréciation de l'administration fiscale. Quel est l'avis de

qui pourrait faire l'objet de discussions, mais à un constat de l'éligibilité, ou non, d'un organisme au régime du mécénat. Il n'est donc pas nécessaire d'allonger particulièrement ces délais, d'autant qu'une association pourrait

M. le président

à ses donateurs. Il s'agit de décisions individuelles, qui résultent d'une analyse propre à la situation de chaque organisme. Un tiers des rescrits rendus chaque année par la DGFiP portent d'ailleurs sur le mécénat. En outre, certaines de ces décisions peuvent apporter un éclairage sur un point de droit

fait pour une raison très simple : les services du ministère de l'économie et des finances nous ont indiqué dans l'oreillette qu'ils n'avaient aucun moyen ! La meilleure façon de constater qu'on est en train d'installer une usine à gaz

M. Sébastien Meurant. Afin de garantir le respect des principes de la République, les associations de financement électorales ou mandataires financiers doivent répondre aux mêmes conditions que les autres associations délivrant des reçus fiscaux. Cela permettrait un axe de contrôle de toute volonté de politique électoraliste séparatiste. Quel est l'avis de

soumis à un contrôle financier distinct qui dépend, non de l'administration fiscale, mais de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). À ce titre, ils sont déjà soumis, en application de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique,

émettent des documents alléchants, promettant une déduction d'impôt, pour des objets absolument contraires à l'ordre public français. Le ministère de l'économie et des finances nous a expliqué qu'il n'avait pas les moyens de suivre de tels dossiers et qu'il revenait au ministère de l'intérieur, chargé des

Comme le souligne le juriste Jean Rivero, « Les textes législatifs, les rapports parlementaires qui les commentent, les circulaires qui ont accompagné leur mise en application ont toujours entendu la laïcité en un seul et même sens, celui de la neutralité religieuse de l'État. thèse de doctorat sur la pensée religieuse et l'impôt, affirme sans ambiguïté que, du point de vue fiscal, « cette neutralité présente la forme de l'absence de prise en compte de la confession du contribuable dans le traitement de ses dettes fiscales ». en mettant fin au financement indirect des cultes, car la réduction d'impôt pour les dons s'apparente bien à une prise en charge par l'État de la dépense du contribuable. Pour prendre un exemple concret, quand un ou une fidèle souhaite donner 100 euros à un culte, il fait assumer un coût de 66 euros à l'ensemble de la collectivité. L'instauration d'un plafond de revenu imposable concerne l'ensemble des dons relevant de l'article 200 du code général des impôts et constitue donc une mise en concurrence entre les différentes causes bénéficiant d'une réduction fiscale. Ainsi, comme le souligne l'auteur précité, les contribuables peuvent arbitrer entre plusieurs affectations, les unes relevant de l'intérêt général- les organismes ayant un caractère éducatif, social, humanitaire ou encore sportif -et les associations cultuelles, c'est-à-dire privées, car les activités religieuses sont considérées comme relevant de la Enfin, on peut souligner le caractère doublement inégalitaire de la fiscalité des dons aux associations cultuelles. D'une part, celle-ci ne concerne que les contribuables imposables au titre de l'impôt sur le revenu, les croyants qui font partie de la moitié la plus pauvre de la population étant priés de payer leurs dons eux-mêmes ; d'autre part, la subvention publique est d'autant plus élevée que le croyant a les moyens de faire un don important, jusqu'à 20 % de son revenu. Il convient donc de faire cesser immédiatement cette interposition de l'État entre un culte et ses fidèles.

En outre, supprimer ces avantages fiscaux à un moment où l'on souhaite que les associations cultuelles n'aillent pas chercher leur financement ailleurs

la collectivité publique en assume 66 euros, vous m'expliquerez la nature de l'équilibre ! En outre trouve-t-on juste que ceux qui sont imposés sur le revenu et qui font ce type de dons puissent être défiscalisés jusqu'à 20 % de la somme, ceux qui sont moins fortunés, qui ont moins de revenus, mais qui souhaitent participer au financement d'un culte, n'ont pas ce droit ? J'avoue avoir du mal à comprendre l'équilibre dont

amendement tend à supprimer l'exonération sur les dons et les legs. Selon une étude de la Fondation de France en 2015, le total de la générosité reçue par l'Église catholique à travers les paroisses et les diocèses s'élève à 630 millions d'euros en 2015, dont environ 40 % font potentiellement l'objet de déductions fiscales. L'État se serait donc privé de 252 millions d'euros pour cette seule année, au profit d'un culte. Les dons et legs représentent 100 millions d'euros de cette somme. Là encore, à l'instar des dons, ce financement indirect des cultes donne lieu à une concurrence entre différentes institutions et nuit, notamment, aux libéralités à destination des organismes publics. Ainsi, les libéralités consenties à l'Église en 2015 sont, pour la même nature, vingt fois supérieures à la somme perçue par l'État, presque deux fois supérieures à l'intégralité des dons et legs reçus par ses opérateurs et deux fois supérieures à ce que perçoivent les collectivités territoriales. En résumé, la seule Église catholique recueille autant de dons et de legs que tous les acteurs publics confondus. Si vous estimez que l'État, ses opérateurs et les collectivités territoriales sont suffisamment bien dotés et que les dons et legs ne

qui a accueilli près de 12 000 patients pendant l'année 2019. Au-delà de 30 euros versés chaque année pour les associations cultuelles par chacun des 50 millions d'adultes résidant en France, il est impératif de revenir à un modèle de financement sans exonération fiscale sur les donations et legs pour que l'État et le Gouvernement sortent enfin de cette ambiguïté coupable quant au financement des cultes.

Benbassa, sur l'article. Cet article concerne la suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif en cas de condamnation pénale.

En effet, depuis 1993, la loi sanctionne les actions empêchant l'accès à l'information sur l'interruption volontaire de grossesse, en ôtant à certains organismes sans but lucratif leurs avantages fiscaux. Devons-nous rappeler à cette assemblée que l'accès à l'information sur l'IVG est une nécessité de santé publique ? La question de l'avortement concerne évidemment toutes les classes sociales, mais ce sont particulièrement les femmes les plus précarisées financièrement qui ont recours à cette pratique, comme le montrent les chiffres du planning familial.

pas été convaincu par les arguments qui ont conduit à opérer cette modification. Aujourd'hui, la liste des infractions susceptibles d'entraîner la suspension des avantages fiscaux prévus par le texte initial de l'article 12 ne comprend que des manquements de nature économique ou faisant peser une menace grave sur la société : terrorisme apologie du terrorisme, etc. On considère donc que le délit d'entrave à l'IVG ne pourrait pas s'inscrire dans cette logique,